Monsieur le président,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

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j'ai le profond regret de vous faire part du décès, survenu cette nuit, de notre collègue Patrick Boré, qui était sénateur des Bouches-du-Rhône depuis août 2020. M. le président du Sénat prononcera son éloge funèbre ultérieurement, mais je tiens d'ores et déjà à saluer sa mémoire.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de présenter une nouvelle fois à la Haute Assemblée le projet de révision constitutionnelle complétant l'article 1 de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement. La genèse de cette réforme historique en faveur du climat, de l'environnement et de la diversité biologique est connue de tous ; je me bornerai donc à rappeler que le projet qui vous est soumis est d'abord le fruit du travail et de l'engagement des 150 Français de la Convention citoyenne pour le climat. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Ce projet tient aussi à l'engagement du Président de la République de reprendre leur proposition citoyenne de modification de l'article 1 de la Constitution, dans le cadre d'un projet de loi constitutionnelle. Nos précédents débats avaient fait apparaître que les désaccords se cristallisaient sur l'emploi de deux des dix-huit mots du projet de loi. Ces deux mots, qui ont donné lieu à de savantes exégèses, sont les verbes « garantir » et « lutter ». Vous le savez, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont souhaité, dans un esprit d'ouverture et de conciliation,

Je comprends, au regard du projet proposé par votre commission et qui fait l'objet d'un amendement de réécriture de l'article unique, que la main tendue n'a pas été saisie. Je le regrette, car vous fermez ainsi la possibilité pour les Français de s'exprimer sur le sujet de première importance qu'est l'avenir écologique de notre pays. Au soutien de la proposition de réécriture, vous avez reproché au Gouvernement d'entretenir zones d'ombre et contradictions quant aux effets juridiques attendus du projet de révision constitutionnelle. Je vais donc m'employer, une nouvelle fois, à préciser le sens et la portée de cette réforme. Je dirai quelques mots, pour commencer, sur le texte que vous proposez. Vous souhaitez indiquer que « la France agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004 On peut se demander, à la lueur de cette rédaction bien timide, si ce qui vous inquiète, finalement, ne réside pas tant dans les prétendues incertitudes juridiques entourant notre projet volonté, pleinement assumée par la majorité présidentielle, de renforcer juridiquement la préservation de l'environnement. À l'inverse, la rédaction que vous proposez ne produirait aucun effet juridique nouveau, comme votre commission l'a d'ailleurs reconnu. À l'heure où nous vivons une crise climatique majeure qui inquiète les Français et mobilise, en particulier, notre jeunesse, première concernée par les conséquences de cette crise, une réforme purement symbolique n'est pourtant pas envisageable. Il n'est pas possible de convoquer les Français à un référendum pour leur dire : Nous réformons la Constitution, mais notre but est de ne strictement rien changer ». Or c'est cela que vous nous proposez, ne rien changer en répétant le préambule de notre Constitution et en renvoyant simplement à la Charte de l'environnement, qui existe déjà. Le Gouvernement et l'Assemblée nationale pensent au contraire qu'il faut assumer pleinement la responsabilité historique qui est aujourd'hui la nôtre et affirmer que la portée juridique de la protection de l'environnement doit évoluer, que ce qui est une ambition doit devenir une garantie. Je souhaiterais tellement vous convaincre du bien-fondé du projet repris de la Constitution citoyenne pour le climat ! Il s'agit, tout d'abord, de rehausser la protection de l'environnement au coeur de nos principes constitutionnels. Certes, comme vous le savez, elle est inscrite dans la Charte de l'environnement résultant de la loi constitutionnelle du 1 mars 2005. Cette Charte, mentionnée dans le préambule de notre Constitution, fait donc pleinement partie du bloc de constitutionnalité, et le Conseil constitutionnel, par sa jurisprudence récente, en particulier par deux décisions de 2020, a contribué à renforcer les principes qu'elle contient. Il subsiste toutefois d'importantes limites. En effet, dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que la préservation de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constituait seulement un objectif à valeur constitutionnelle. Je rappelle qu'un objectif à valeur constitutionnelle, à la différence d'une règle constitutionnelle ayant un caractère impératif, n'emporte qu'une obligation de moyens et nécessite, pour sa mise en oeuvre, l'intervention du législateur. Nous voulons ici mettre en place un principe à valeur constitutionnelle, qui pourra être invoqué même lorsque le législateur n'est pas intervenu. Par ailleurs, je vous rappelle que les objectifs à valeur constitutionnelle ne sont théoriquement pas invocables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il s'agit donc bien de renforcer le poids constitutionnel de la protection de l'environnement. Ensuite, le Gouvernement vise, avec ce projet, à instaurer un véritable principe d'action des pouvoirs publics, nationaux comme locaux, en faveur de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique. Bien sûr, l'article 2 de la Charte prévoit déjà pour toute personne le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Mais, ici, nous allons plus loin : nous voulons créer, à la charge des pouvoirs publics, une garantie de la préservation de l'environnement.

fasse l'objet d'un tel rejet de la part de votre Haute Assemblée : faut-il de nouveau rappeler que notre Constitution l'emploie déjà ? Ainsi, lorsque les constituants ont inscrit dans la Constitution, en 1946, la garantie de la santé et de la protection matérielle, du repos, des loisirs, ils n'ont pas imposé une responsabilité automatique de l'État pour toute personne malade ou en grande précarité. Les dangers que vous dénoncez, sur ce point, sont illusoires. S'agissant des effets juridiques du verbe « garantir » sur la mise en jeu de la responsabilité des personnes publiques, je ne puis que répéter ce qui a déjà été exposé : il est certain que l'État peut déjà voir sa responsabilité engagée en matière environnementale, mais nous voulons aller plus loin et créer une quasi-obligation de résultat ou, comme je l'ai toujours dit, une obligation de moyens renforcée pour les pouvoirs publics. Cela signifie tout simplement faciliter la charge de la preuve pour les requérants et, à l'inverse, rendre beaucoup plus difficile pour la personne publique mise en cause de s'exonérer de ses obligations. Il ne s'agit donc pas de se satisfaire des carences ou de l'inaction des pouvoirs publics pour les condamner ensuite, mais bien au contraire de les obliger à agir pour protéger concrètement et efficacement l'environnement. La Constitution doit s'adapter aux enjeux et aux défis de notre temps. Elle doit donc être aujourd'hui à la hauteur du défi écologique majeur auquel notre pays se trouve confronté. Voilà pourquoi le Gouvernement et l'Assemblée nationale, à l'unisson de la Convention citoyenne pour le climat, entendent garantir la protection de l'environnement. Ce combat est aujourd'hui le nôtre, il devrait aussi être le vôtre, car c'est le combat de la France pour le siècle à venir.

nous pouvons le comprendre, mais tout de même : il ne suffit pas que les gouvernements affirment quelque chose pour que cela soit la vérité ! Très bien ! Le travail

mais dont il nous revient à nous, parlementaires et constitutionnalistes pour la circonstance, d'apprécier la réalité des effets. Nous avons toujours dit à cette tribune que nous souhaitions naturellement que les parlementaires

Le Sénat est donc saisi, en deuxième lecture, d'un projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1 de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 11 mai dernier. La commission des lois n'a pu que constater, à regret, que les conditions d'un accord entre les deux assemblées sont encore très loin d'être réunies. Je vous rappelle que le projet initial du Gouvernement, décalque de l'une des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, prévoyait d'insérer à l'article 1 de notre Constitution une phrase selon laquelle la France « garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Il avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sans modification. Saisi de ce texte, le Sénat avait observé que la rédaction proposée avait une portée juridique beaucoup trop vague pour pouvoir être adoptée en l'état. Comme le soulignait alors la commission, et contrairement aux allégations qui ont été exprimées, les pouvoirs publics sont d'ores et déjà soumis à de fortes obligations de valeur constitutionnelle ayant pour objet la protection de l'environnement, obligations qui découlent de la Charte de l'environnement de 2004. En revanche, compte tenu, notamment, de l'emploi du verbe « garantir » et du défaut d'articulation avec la Charte, il avait paru impossible à notre commission de déterminer avec un tant soit peu de précision les effets des dispositions envisagées, d'une part, sur l'engagement de la responsabilité des personnes publiques, et, d'autre part, sur la validité des actes des pouvoirs publics. Le Sénat avait donc substitué aux dispositions proposées une phrase selon laquelle la France « préserve l'environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004 ». Cette rédaction supprimait la référence à la notion de « garantie » et levait, grâce à un renvoi exprès, tout problème d'articulation entre l'article 1 de la Constitution, modifié, et la Charte de l'environnement, partie intégrante du bloc de constitutionnalité. La substitution du verbe « agir » au verbe « lutter », déjà suggérée par le Conseil d'État, visait seulement, quant à elle, à éviter un effet rhétorique dénué de toute portée juridique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sous couleur de rechercher un terrain de compromis avec le Sénat, a presque intégralement rétabli le texte initial, en acceptant seulement le remplacement du verbe « lutter » par le verbe « agir »,

Les députés n'ont pas cherché à répondre aux arguments juridiques exposés par le Sénat. Bien au contraire, les débats en deuxième lecture à l'Assemblée nationale n'ont fait qu'entretenir le flou sur les effets que le Gouvernement et sa majorité Permettez-moi d'en citer quelques exemples. Le Gouvernement, après avoir répété à qui voulait l'entendre que son texte visait à instituer « un véritable principe d'action des pouvoirs publics » en faveur de la protection de l'environnement, a enfin reconnu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale que la Charte de l'environnement s'applique aux autorités publiques depuis seize ans. C'est une avancée que nous relevons. Alors qu'il prétendait auparavant que le projet de révision visait à assigner aux pouvoirs publics une « quasi-obligation de résultat » en matière de protection de l'environnement, le Gouvernement ne parle plus désormais que d'une « obligation de moyens renforcée

les pouvoirs publics, si leur responsabilité est recherchée en justice, à établir eux-mêmes la démonstration qu'ils ont accompli toutes les diligences raisonnables pour assurer la préservation de l'environnement. Soit, mais il faut tout de même beaucoup d'imagination pour faire produire au verbe « garantir » de tels effets sur le régime de la preuve dans le procès administratif. La notion de garantie, dans le langage courant comme dans le langage juridique, a une autre signification. Pendant ce temps, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale prétend toujours que le texte aurait pour effet « d'ériger la protection de l'environnement en principe constitutionnel »,

Il a également déclaré que le texte adopté par les députés pourrait constituer « le support d'actions en carence contre le législateur », ce qui, pour le coup, constituerait une nouveauté, puisque, dans notre État de droit et conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, aucune juridiction n'a le pouvoir d'adresser des injonctions au législateur non plus d'ailleurs que de condamner l'État à réparer les dommages causés par d'éventuelles carences du législateur. Il est bien évident que la disposition proposée ne suffirait pas, à elle seule, à opérer un tel bouleversement juridique. Si l'on en croit les déclarations faites en séance publique par le rapporteur de l'Assemblée nationale, la prétendue concession faite au Sénat serait l'expression de « l'esprit de dépassement et de rassemblement » qui, comme chacun sait, anime le parti majoritaire ... Au moins, cela ne manque pas d'humour.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, pour la seconde fois, nous sommes convoqués pour débattre du projet de loi constitutionnelle visant à modifier l'article 1 pour y inscrire la protection de l'environnement. Sans surprise, le Sénat, en première lecture, a réécrit le texte afin d'en affaiblir la portée, réduisant l'insertion à une sorte de tautologie renvoyant à la Charte de l'environnement.

Nous voilà donc coincés dans un débat purement sémantique sur la portée concrète des verbes « garantir », « préserver » et « agir », dans le cadre d'une navette qui pourrait se poursuivre éternellement. J'avais dit, en première lecture, que nous nous inscrivions en faux contre cette instrumentalisation du Parlement, une manoeuvre dilatoire aux effets pervers. En effet, loin de consacrer constitutionnellement la protection de l'environnement, ces rédactions fragilisent au contraire la Charte, sans créer aucune obligation de quasi-résultats, malgré vos déclarations, monsieur le garde des sceaux. Pour cette raison, nous vous avions proposé de réduire ces modifications constitutionnelles, non pas aux symboles, mais à l'enrichissement de la Charte, selon les principes de solidarité écologique et de non-régression. Ces dispositions utiles auraient permis au juge constitutionnel de censurer un certain nombre de lois récentes, comme la réautorisation des néonicotinoïdes ou les ASAP. Les faits sont cependant têtus, et l'objectif du Gouvernement, comme de la majorité sénatoriale, n'est pas d'être utile, mais bien de faire illusion. Je dois vous le dire : cette farce constitutionnelle commence

Pour bien me faire comprendre, je citerai de Visconti et son fameux « il faut que tout change pour que rien de change », qui décrit exactement la stratégie de ce gouvernement en matière de transition écologique, avec la complicité de la majorité sénatoriale. Non ! La discussion du projet de loi portant Nous avons passé deux semaines à débattre d'une poignée de mesures insignifiantes, déjà obsolètes, qui ne remettent en cause ni l'organisation du système financier et de production ni la préservation des intérêts économiques et les droits acquis. Cette manière de procéder décrédibilise le Parlement et la politique dans son ensemble.

Cette réforme constitutionnelle passe ainsi à côté de l'essentiel : elle ne porte pas les évolutions constitutionnelles dont notre pays a tant besoin pour sortir de la présidentialisation du régime, pour engager l'irruption citoyenne et le respect de la souveraineté populaire, notamment en rééquilibrant les pouvoirs en faveur du Parlement. Parlement. Concernant le climat, aucune réforme constitutionnelle n'aura d'effectivité sans mettre en oeuvre de politiques publiques ambitieuses. Il faudrait ainsi, et prioritairement, faire respecter la Charte. Il faudrait également remettre en cause les accords de libre-échange et les politiques libérales de privatisation et de casse du service public ; engager un vaste plan de reconquête dans les secteurs clés que sont les transports et l'énergie, en s'appuyant sur les opérateurs publics, EDF et la SNCF, voire en revenant dans le capital de certains opérateurs ; enfin, respecter les engagements contractés dans l'accord de Paris. Des décisions de justice administrative récentes nous y obligent. Le Conseil d'État vient ainsi d'enjoindre le Gouvernement, dans le cadre de « l'affaire du siècle », à prendre toutes les mesures utiles pour que la France tienne ses objectifs. Dans un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris avait déjà reconnu une carence partielle de l'État, qui engageait sa responsabilité. Pour reprendre l'image de la maison qui brûle, je dirais que depuis le début de ce mandat, c'est à grand renfort d'essence que vous nous nourrissez ce feu. Il ne restera bientôt que des cendres et la colère de nos concitoyens ; une colère légitime face à l'inaction climatique de la France, mais aussi, et surtout, face à l'incapacité du politique à agir pour garantir à chacun des conditions d'existence dignes, trop occupés que vous êtes à démanteler tous les conquis sociaux. Nous confirmons donc notre vote négatif sur ce projet de loi inutile et inopérant, qui n'a d'autre objet que détourner notre attention des véritables objectifs de ce gouvernement. La parole

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'Assemblée nationale et le Gouvernement n'ont pas souhaité donner suite

le Sénat. Le premier concerne l'incertitude béante quant aux conséquences d'une telle garantie par la Nation. Je veux bien admettre que, sur ce point, le choix du verbe ait une incidence. Deux autres points

Où est la volonté de dialogue ? Où est le désir d'aboutir à un accord ? Par ailleurs, vous nous dites que les propositions du Sénat

la Cour de cassation a pu vous poser quelques problèmes, monsieur le garde des sceaux, sur la notion de décence en matière de détention, c'est parce qu'il y a eu des dispositions

que la volonté de dialogue exprimée par le Sénat n'a pas été saisie par l'Assemblée nationale. Par conséquent, le groupe Union Centriste ne manquera pas d'approuver la proposition faite par la commission des lois. La parole est

si j'étais taquin, je dirais que tout cela devient croquignolesque, alors que le sujet appelle gravité et sérieux. Comme dans un parlementaire d'j'ai le sentiment que nous sommes enfermés dans une boucle temporelle. De nouveau, nous voilà débattant d'une révision constitutionnelle portant sur l'article 1 de notre Constitution, sans que la navette parlementaire ait permis d'avancer. De nouveau, cette révision donne à lieu à des débats de pharisiens dans lesquels chacun, Gouvernement, majorité à l'Assemblée nationale et majorité au Sénat, feint de chercher un compromis dans un jeu de de poker menteur. Ces postures parlementaires et gouvernementales font peser un doute sérieux sur l'organisation d'un référendum ou la tenue d'un Congrès avant la fin du quinquennat. Dès l'origine, il y avait d'ailleurs peu de chances d'aboutir, au regard des délais, ce qui révèle l'insincérité de la volonté initiale de l'exécutif dans cette entreprise. Bref, « tout ça pour ça ». Aussi, mes chers collègues, quel est le sens de notre discussion ? La loi La loi fondamentale et la préservation de la planète méritent-elles autant d'instrumentalisation politique, au point de perdre de vue l'essentiel de ce qui devrait nous occuper ? Nul, ici ou ailleurs, n'a besoin du décryptage du jeu de dupes qui se joue.

Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, ce texte relève purement du prétexte. Emmanuel Macron cherche à déporter une double responsabilité sur le Sénat et, singulièrement, sur la majorité sénatoriale.

s'agit de la responsabilité de ne pas honorer l'engagement pris devant la Convention citoyenne pour le climat, permettant ainsi au Président de la République de s'en dédouaner. La majorité sénatoriale, quant à elle, tente d'échapper à ce piège politique grossier tendu par le Président de la République. Elle est face à un dilemme : faut-il offrir un référendum au chef de l'État à la veille de la présidentielle de 2022 ou faut-il le bloquer, quitte à cultiver le cliché, certes erroné, d'une chambre ringarde en décalage avec son temps ? La majorité sénatoriale a choisi : elle préfère endosser le blâme de ne pas réviser la Constitution, tout en dénonçant l'Assemblée nationale. Ainsi, s'appuyant sur l'avis du Conseil d'État et la responsabilité du constituant, elle invoque une rédaction juridique incertaine, qui ferait peser des risques sur notre ordre constitutionnel. Elle lui préfère une rédaction dont elle reconnaît la faible portée normative, sans méconnaître sa portée symbolique, mais en la réduisant à un placebo. Malheureusement, ces discussions sémantiques, aussi intéressantes qu'interminables, se tiennent au détriment de la finalité. En définitive, la majorité sénatoriale fait ce que l'exécutif attendait d'elle et vient ripoliner en vert l'image d'Emmanuel Macron. Dans une des matinales radios d'aujourd'hui, le porte-parole du Gouvernement, connu pour sa hauteur de vue, son sens de la mesure et sa sincérité, parlait du Sénat qui empêcherait de lancer le référendum et dont la majorité ne serait généralement pas favorable aux mesures en faveur de l'environnement, par climatosceptisme ... Fermez le ban Las, pendant que chaque joueur d'échecs tente de mesurer le coût politique de telle ou telle option, quel est le résultat de ce manège ? Quel est le coût pour la démocratie et pour l'avenir de la planète ? Telles sont les vraies questions que nous devrions nous poser, c'est-à-dire celle du fond, et non de la forme. Du point de vue démocratique, tout d'abord, je crains que nos débats parlementaires suscitent plus de désintérêt qu'autre chose de la part des Français que nous avons pour responsabilité de représenter. Les calculs politiques des uns ne font qu'alimenter la crise démocratique aux yeux des autres ; à cet égard, n'oublions pas le coup de semonce du dernier scrutin électoral. Du point de vue démocratique encore, on peut contester la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat et considérer que ce ne sont pas 150 citoyens, pourtant impliqués, qui devraient indiquer la marche à suivre au Parlement.

assume son travail de législateur. Du point de vue de la planète, ensuite, la transition écologique se retrouve l'otage de considérations politiques qui n'ont rien à voir avec elle. Parlementaires et juristes, nous avons disserté à l'envi sur les verbes « agir » et « garantir », au détriment de l'enjeu final.

Pourtant, avons-nous une responsabilité en matière de réchauffement climatique ? Qui, dans cet hémicycle, peut oser répondre par la négative à cette question ? Qui peut oser s'affranchir d'une quelconque responsabilité envers les générations futures ? sur l'évolution du climat, le GIEC, les rapports se suivent et se ressemblent, s'accumulent, s'entassent et se répètent sans jamais se contredire : la situation n'est plus tenable, et la crise sanitaire en est l'une des illustrations. Le prérapport du GIEC indique qu'une augmentation du réchauffement climatique au-delà de 1,5 degré pourrait déjà entraîner « des conséquences graves, pendant des siècles, et parfois irréversibles ». L'organisation météorologique mondiale estime à 40 % la probabilité de dépasser ce seuil d'ici à 2025. Pour ceux qui préfèrent le droit- ils sont nombreux ici -, la lecture de la récente décision du Conseil d'État est éclairante : celui-ci a sommé l'État d'agir pour le climat en donnant au Gouvernement jusqu'au mois d'avril 2022 pour prendre « toutes les mesures utiles », afin d'atteindre ses objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre, sous peine d'astreinte financière- une future décision qui interviendra donc en pleine campagne présidentielle. Pour les contemplatifs- il y en a quelques-uns -, l'actualité parle d'elle-même : vagues de sécheresse, inondations à répétition, phénomènes de submersion,

Notre Charte de l'environnement n'est pas suffisante. La Constitution doit donc s'adapter aux nécessités de notre temps. Deux questions éminemment politiques auraient dû animer notre débat et nos décisions.

Dans cette perspective, nous étions attachés à l'intégration de la notion complémentaire de « préservation des biens communs mondiaux », qui nous semblait centrale et qui a fait l'objet d'une proposition de loi socialiste forte, portée par notre collègue Nicole Bonnefoy. Le droit de propriété doit pouvoir être contraint pour préserver ces biens communs. C'était d'ailleurs l'esprit de l'un des projets de texte constitutionnel pour la IV République, projet qui n'a pas été retenu.

si le vote conforme est désormais plus que compromis, nous ne souhaitons pas ajouter de l'obstruction à l'obstruction. Nous avons préféré ne pas déposer d'amendement et voter contre ceux de la majorité. La parole

Des effets météorologiques violents sont répertoriés à intervalles très réguliers ; la France les a subis en nombre cette année : ils ont des impacts sur tous nos concitoyens, dans leur vie, mais aussi dans leur travail. Je pense notamment à nos agriculteurs, qui vivent encore les conséquences du gel du début du printemps Sur mon territoire, nous vivons, depuis une vingtaine d'années, une sécheresse toujours plus précoce et grave, ainsi que des saisons de moins en moins prévisibles. Plus personne ne nie aujourd'hui ces changements, que nous cherchons à enrayer. Le projet Le projet de loi constitutionnelle, que nous retrouvons dans cet hémicycle en deuxième lecture, a encadré l'étude d'un autre projet, celui du projet de loi Climat et résilience. Les centaines d'articles qu'il contient concernent des domaines très variés, ayant pour objectif principal la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre dans un avenir très proche. Le Sénat a travaillé à insérer ce texte dans une logique réaliste et pragmatique. Nous ne pouvons pas orienter notre pays avec la seule logique environnementale. Notre transition, pour être efficace, doit être ancrée dans le réel. L'article unique dont nous faisons une nouvelle étude est arrivé de l'Assemblée nationale avec des termes encore différents de ceux que nous avions modifiés lors de notre première lecture. L'examen que nous en avons fait la semaine dernière en commission des lois soulève presque les mêmes problèmes qu'à l'origine.

La vision du groupe Les Indépendants reste la même qu'en première lecture : nous ne pouvons faire entrer l'incertitude dans notre Constitution. S'il y a une urgence, c'est surtout celle de faire les choses bien.

La protection de l'environnement impliquera inévitablement les volets sociaux et économiques de notre système. Une écologie humaniste et libérale fera de nos investissements et de nos innovations autant de moteurs primordiaux de la lutte contre le changement climatique. Demain, nous circulerons dans des transports propres, ce qui représente l'un de nos plus grands défis. Nous aurons décarboné des pans entiers de nos industries les plus polluantes, comme celles de l'acier ou du ciment, très émettrices de CO2. Notre économie sera beaucoup plus circulaire. Nos bâtiments, tout au long de leur vie, nous permettront des économies d'énergie. Le numérique, qui prend une place grandissante dans nos habitudes, sera également moins énergivore. Notre mode de vie aura évolué et sera beaucoup plus respectueux. cela ne se fera que si l'on s'en donne la possibilité et si notre relance et notre croissance sont vertes. Cela ne se produira que si la protection de l'environnement est pensée dans son ensemble, avec tous les acteurs et citoyens, pas seulement français, mais du monde entier. Pour cela, notre Constitution doit rester une alliée. Nous ne sommes pas contre le fait d'inscrire la préservation de notre environnement dans son article 1. Nous souhaitons simplement le faire efficacement en en mesurant toutes les conséquences. Il faut écarter le flou autour de la définition future du verbe « garantir ». Il faut également se préserver d'un potentiel glissement vers un gouvernement des juges. Je le répète, les arbitrages éminemment politiques ne peuvent être confiés aux juges. Ces arbitrages doivent rester le lieu de discussion des élus.

et sommes même heureux de les accepter. La France doit donc « agir pour lutter contre le changement climatique et en faveur de la préservation de l'environnement et de la diversité biologique ». Elle doit le faire dans les conditions que la Charte de l'environnement nous propose. Cette Charte, qui fait de la protection de l'environnement un objectif de valeur constitutionnelle, est un trésor de notre bloc de constitutionnalité sur lequel nous avons la chance de pouvoir nous appuyer. Ne l'oublions pas. est le sens de la rédaction que propose notre rapporteur, un amendement dont nous allons discuter. Sous réserve de l'adoption de cet amendement, dont je ne doute pas, le groupe Les Indépendants votera à l'unanimité en faveur de ce texte, dans sa rédaction modifiée.

grâce à l'action conjuguée du Président de la République et de son gouvernement et de la majorité de droite du Sénat. « La vie sur terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas.

Nous n'avons plus le temps de tergiverser. Je refuse de me résigner à une inaction de notre pays ou, comme l'a encore rappelé le Conseil d'État jeudi dernier, à une action bien trop peu ambitieuse. Je le rappelle devant cette assemblée parfois trop frileuse vis-à-vis des mécanismes de démocratie participative, la Convention citoyenne pour le climat a émis, dans ses travaux, le souhait d'inscrire le principe de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique au sein de l'article 1 de notre Constitution. Soyons clairs, le texte initial du Gouvernement et celui qui nous revient de l'Assemblée nationale ont des limites. Notre groupe le sait, le dit et le montre au travers des amendements que nous avons déposés. Nous aurions préféré une rédaction différente, plus complète, demandée depuis des années par tout le mouvement écologiste.

Vous n'hésitez pas à affirmer que nous sommes en danger et qu'il faut sauver la vie sur terre. Mais vous renâclez à l'idée que ce combat soit essentiel et que nous puissions utiliser tous les moyens pour le mener. Pourtant, partout sur le terrain, nos élus et nos concitoyens ont compris et mettent en oeuvre, eux, prioritairement, des mesures et des actions dans ce sens.

Aussi, inscrire cette garantie au coeur de l'article 1 pourrait devenir un outil majeur pour définir les contours de traités commerciaux internationaux acceptables pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Je vous l'ai déjà dit, mes chers collègues, je crains que votre posture ne soit politique, et en rien technique. Ce jeu de dupes a certes été lancé par le président Macron et son gouvernement, mais vous acceptez bien volontiers d'y jouer, vous appuyant l'un sur l'autre et faisant fi de la réalité de l'urgence. Vous souhaitez tous, à un an de l'élection présidentielle, vous rejeter la faute de la non-tenue d'un référendum. Il est évident que les seuls qui avancent de manière transparente sur le sujet, depuis longtemps, sont les écologistes, que nous représentons ici. L'urgence climatique nous guide. Nous souhaitons que, à l'avenir, les exécutifs au pouvoir ne puissent ignorer la protection de l'environnement dans leur action. L'alternance politique de notre pays ne saurait se faire au détriment de l'écologie, donc des citoyens. Osons Osons présenter ce projet à l'ensemble des citoyens ; n'ayons pas peur d'eux. Notre ambition de voter ce texte dans les mêmes termes que ceux de l'Assemblée nationale est ancrée dans notre devoir envers les citoyens, afin de leur permettre de débattre, de se prononcer et d'être consultés. Ce projet de loi constitutionnel n'est sûrement pas à la hauteur des enjeux, tout comme le projet de loi Climat et résilience ne l'a pas été. Néanmoins, il peut et il doit constituer une étape essentielle vers une prise en compte meilleure et plus systématique des enjeux environnementaux. Bien sûr, les renoncements successifs de ce gouvernement sur les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, sur l'utilisation du glyphosate, sur le retour de l'utilisation des néonicotinoïdes et sur tant d'autres ne seraient pas absous par ce semblant de virage écologique. Nous ne sommes pas dupes de l'ambition du Gouvernement d'utiliser le soutien à ce texte comme un faire-valoir d'une politique environnementale lacunaire. Cependant, nous devons avancer. La Convention citoyenne pour le climat, les marcheurs pour le climat, les collectifs et associations écologistes, les scientifiques et experts et les citoyens qui agissent quotidiennement nous le demandent. Même si ce texte ne va pas au bout de la démarche que les écologistes portent depuis des années, il est temps d'agir plus vite et plus fort. Nous sommes prêts à voter ce texte dans sa version issue de l'Assemblée nationale. Nous voterons, bien entendu, contre les amendements

ce deuxième rendez-vous sur le projet de loi constitutionnel visant à inscrire la préservation de l'environnement à l'article 1 de notre Constitution nous amène à un double constat. D'une part, contrairement à ce qui avait été auguré ici ou là lors de l'examen en première lecture, la navette a bien suivi son cours. D'autre part, la politique des petits pas, que traduisent les modifications portées par les rapporteurs des deux assemblées, ne suffit pas à poser les bases d'un compromis. La deuxième lecture, telle qu'elle se profile, confirme en l'état les vives réticences de la majorité sénatoriale sur la révision proposée par la Convention citoyenne pour le climat et reprise par l'exécutif dans la perspective d'une adoption par référendum. Nous le regrettons. Alors que nous pouvons tous partager la conviction que la France doit s'armer de nouveaux instruments juridiques pour répondre à l'urgence climatique, la divergence de méthode persiste. persiste. Elle s'est focalisée, dans nos débats, sur la portée des termes retenus dans le projet de révision, mais elle traduit je crois, au-delà de la seule sémantique, une différence d'ambition intrinsèque. lors de l'examen du texte en première lecture, nous nous étonnions qu'une partie de l'hémicycle défendît l'adoption d'une réécriture du rapporteur qui revendiquait l'absence d'effet juridique. La réécriture de substitution qui nous sera présentée ultérieurement par le rapporteur et le président du groupe Les Républicains semble confirmer cette volonté de priver d'effet juridique la révision constitutionnelle. Le renvoi tautologique à la Charte de l'environnement en témoigne. Notre étonnement ne peut qu'être affermi à l'examen du rapport de deuxième lecture, qui se borne à déconstruire les conséquences du texte adopté par l'Assemblée nationale, sans évoquer les effets recherchés par la rédaction alternative proposée. Certes, l'absence de consensus entre les constitutionnalistes sur la portée des différents verbes retenus ne concourt pas à clarifier le débat. Elle nous enjoint en tout cas au parti pris. La révision portée par le Gouvernement serait tantôt inutile, tantôt dangereuse. Dans la mesure où il nous semble difficile de considérer qu'un texte puisse être à la fois dépourvu d'effet et porteur d'une menace, nous choisissons la voie médiane. La portée de ce texte était déjà précisée dans les travaux préparatoires de l'Assemblée nationale : il ne s'agit pas d'introduire une prééminence de l'environnement sur les autres principes ni de bloquer toute action des pouvoirs publics.

Or les objectifs de développement durable, que nous soutenons, n'ont pas été mis à mal par cette disposition. Mes chers collègues, nous pensons que le texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale ne remet pas en cause le principe d'une conciliation entre les différents droits et libertés fondamentaux.

juridique supplémentaire, dans son appréciation de la constitutionnalité des textes qui lui seront soumis. Il vise, en effet, à renforcer la place de la préservation de l'environnement dans la conciliation du juge. En outre, l'obligation de moyens renforcés mise à la charge des pouvoirs publics accompagne le mouvement jurisprudentiel sur la responsabilité, que l'on a pu observer encore récemment. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, réformer la Constitution n'est jamais un acte anodin. maintenez votre désaccord avec la réforme ambitieuse engagée par la majorité présidentielle, dans la continuité des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et vous nous présentez une proposition de réécriture qui se cristallise encore une fois sur les verbes employés. de nouveau inscrire la révision proposée dans le contexte de la Charte de 2004. Or il ressort des travaux préparatoires du Sénat que cette rédaction ne produira pas d'effet juridique. Si nous poussons le raisonnement à son terme, devons-nous donc comprendre que soutenir le « oui » au référendum consisterait à convaincre les citoyens de se rendre aux urnes pour approuver une révision constitutionnelle dont les auteurs revendiquent qu'elle n'aura pas de portée ? Ce parti pris cynique nous paraît très en deçà de l'urgence environnementale à laquelle nous devons faire face. Le groupe RDPI ne pourra se résoudre à voter le projet de révision constitutionnelle, ainsi réécrit et minoré par la majorité de la Haute Assemblée. La parole est

Elle est la conséquence de l'insuffisance des efforts de l'État en matière environnementale, certes depuis de nombreuses années. Dans le monde, comme dans notre pays, le contentieux climatique n'en est qu'à ses balbutiements. Le verdissement récent de la jurisprudence administrative et constitutionnelle poursuivra son cours, avec ou sans le projet de loi constitutionnelle. Dans son arrêt, le Conseil d'État rappelle que le principe de la protection de l'environnement occupe déjà la plus haute place dans la hiérarchie des normes. inscription à l'article 1 ne lui conférerait donc aucune prééminence d'ordre juridique sur les autres normes constitutionnelles, ce que le Sénat fait mine de craindre. Pourtant, les auditions menées nous ont assez bien éclairés : il n'y aura pas de dérèglement du contentieux, malgré la volonté du Gouvernement de porter un effet accélérateur de l'engagement de la responsabilité pour faute des pouvoirs publics. Le professeur Dominique Rousseau a rappelé qu'il ne fallait pas accorder une valeur juridique plus contraignante aux termes « garantir » ou « préserver », étant donné qu'aucun droit n'est absolu et que le droit constitutionnel ne fait pas la distinction entre une obligation de moyens et une obligation de résultat. Si la réforme devait aboutir, les inquiétudes devraient rapidement se dissiper, du fait du double filtrage en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC, à savoir la saisine indirecte du Conseil constitutionnel par les parties et le contrôle préalable opéré par le Conseil d'État et la Cour de cassation. également que le Conseil constitutionnel, avant de se prononcer, anticipe les incidences économiques, sociales et politiques de ses décisions, et en tient compte. La commission des lois du Sénat choisit donc de maîtriser les conséquences de la réforme pour que celle-ci n'ait très exactement aucun effet, même symbolique. En effet, plus que juridique, cette réforme est d'abord symbolique. Or la Constitution recèle bien des symboles qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit de contester aujourd'hui. Au-delà des symboles, si le Gouvernement voulait nous prouver qu'il entend placer la préservation de l'environnement parmi les priorités de l'action de la France, il pouvait nous le démontrer par des actes, à commencer par un renforcement de l'ambition de la loi Climat. Pour l'instant, tel n'est pas le cas. Certes, le Gouvernement est sans doute allé un peu vite en besogne. L'élaboration de la Charte de l'environnement avait impliqué, quant à elle, la constitution d'un comité d'experts présidé par M. Yves Coppens, et fait l'objet d'assises territoriales. La politique environnementale, au regard du manque d'adhésion d'une grande partie de nos concitoyens, inquiets à juste titre de ses conséquences sociales, méritait que l'on s'y attelle plus longuement. Nous sommes donc pris dans un étau de jeux politiciens qui se concrétisera par une navette infinie. Le citoyen n'est pas dupe, et l'issue de ces débats ne satisfera personne. Ceux qui voudraient aller plus loin dans la préservation de l'environnement estimeront que cette mesure est purement cosmétique. Ceux qui sont d'avis contraire la jugeront dangereuse. Je constate d'ailleurs que, entre la première et la deuxième lecture, le projet de loi constitutionnelle a perdu un certain nombre de voix à l'Assemblée nationale. Pendant que nous nous attardons sur un débat sémantique complètement superfétatoire, le climat, lui, s'emballe. Tergiverser et temporiser nos actions, c'est l'assurance que les restrictions à nos libertés seront, à l'avenir, plus sévères et abruptes. Quant à l'anticipation, elle nous garantit que la transition écologique sera progressive et juste. Or le Haut Conseil pour le climat persiste dans son analyse en raison du retard accumulé par la France, le rythme actuel de réduction annuelle des émissions de CO2 devra pratiquement doubler sur la période du troisième budget carbone, c'est-à-dire entre 2024 et 2028. Nous n'y sommes pas le GIEC, dans son prérapport pour 2022, affirme sans hésiter que l'homme ne survivrait pas à un changement climatique majeur, contrairement à la planète, sans changement radical de ses comportements. Quelle que soit la fin de cette aventure parlementaire, il est plus que certain que la France n'agit pas comme elle le devrait pour la préservation de l'environnement et contre le dérèglement climatique. On peut toujours graver dans le marbre qu'elle agit, serait conforme à la réalité, puisqu'elle le fait malgré tout, mais cette réforme n'apporterait strictement rien si la version proposée par le Sénat devait être retenue. En l'absence de consensus des deux chambres, et lassé par ces manoeuvres comme nous le sommes nous-mêmes, le citoyen se déplacera-t-il si le référendum devait avoir lieu ?

la protection de l'environnement est une exigence constitutionnelle depuis 2005. Aussi, pourquoi pourquoi cette nouvelle réforme constitutionnelle ? Que va-t-elle changer ? Quelles nouvelles obligations implique-t-elle ? Personne, monsieur le garde des sceaux, n'a été capable de le dire, ni la Convention citoyenne pour le climat, ni le Gouvernement, ni même le Conseil d'État, qui a cependant exprimé avec netteté ses réserves.

c'est que l'article 1 de la Constitution n'a pas plus de valeur juridique que la Charte de l'environnement. La distinction entre une règle constitutionnelle et un objectif à valeur constitutionnelle ne dépend pas de la localisation de la norme constitutionnelle dans les textes fondamentaux.

elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Quant à l'article 1, il prévoirait, si ce texte était adopté, que « la République garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique

La garantie de la protection et de la mise en valeur de l'environnement ne serait donc pas corrélée, comme dans la Charte, à l'exigence de conciliation avec le développement économique et le progrès social. Tel est le choix politique qui est opéré. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, monsieur votre projet ne peut pas être sans conséquence. Un troisième élément de certitude tient à ce que la combinaison de l'article 6 de la Charte et du nouvel article 1 sera par conséquent impossible. Ce sera l'un ou l'autre. Et puisque la nouvelle règle fixée à l'article 1 sera la plus récente, elle s'imposera

qui ne mériterait ni un vote du Parlement ni, encore moins, le recours au référendum. Le peuple français ne saurait être convoqué pour ne rien décider. Un référendum ne peut se réduire à une simple opération de communication.

de le dissiper et de nous éclairer sur la portée réelle du texte, vous vous en remettez, en quelque sorte, à la sagesse du Conseil constitutionnel, pour déterminer le contenu le contenu du changement proposé. Cela s'appelle un saut dans l'inconnu. Vous paraissez vous accommoder de cette incongruité. Elle n'a pourtant aucun précédent dans notre histoire constitutionnelle. Elle laisserait le législateur de demain dans l'incertitude et elle placerait les législateurs d'hier et d'aujourd'hui sous la menace de nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité, au résultat tout aussi incertain. Après la deuxième lecture de l'Assemblée nationale, qui en réalité n'a tenu aucun compte de nos travaux, le choix entre les verbes « lutter » et « agir » étant en réalité accessoire s'agissant du réchauffement climatique, nous devrions adopter ce texte comme s'il était à prendre ou à laisser- en somme, à l'aveugle ! Nous devrions renoncer à exercer pleinement notre responsabilité de constituants et accepter ce ce cas singulier d'incompétence constitutionnelle, comme il y a des cas d'incompétence législative, que nulle juridiction ne pourrait évidemment censurer. Cependant, si nous n'avons pas le droit d'adopter une loi floue, à plus forte raison devrions-nous nous interdire de voter une règle constitutionnelle ectoplasmique. Un objectif à valeur constitutionnelle clair, celui de la Charte, vaudra toujours mieux qu'une règle constitutionnelle indéterminée et ambiguë. Cette révision constitutionnelle est à la Constitution ce que les montres de Dali sont à l'horlogerie. Ce pourrait être une nouvelle démonstration de votre sens artistique, monsieur le garde des sceaux, mais, en l'occurrence, votre amour-propre d'auteur ne risque pas d'être frustré, puisque le texte que vous défendez n'est pas le vôtre. est le fruit des réflexions d'un aréopage qui ne s'est pas même donné la peine de vous demander votre avis. Cet aréopage n'a probablement pas pris le temps, non plus, de mettre son expertise juridique au niveau de l'expertise écologique dont il se prévaut.

Cette différence explique sans doute un résultat aussi désolant pour la Constitution que pour l'écologie. Nulle institution de la République, hormis le Sénat, n'a pourtant osé remanier ce projet de loi constitutionnelle, pour lui faire prendre sens et lui apporter la sécurité juridique qui est nécessaire. Il faut remercier le président de la commission des lois, M. Buffet, de s'y être attelé avec l'efficacité et la sagacité que nous lui connaissons. Peut-on imaginer une révision constitutionnelle scellant l'accord du Président de la République, du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat et, en définitive, du peuple français appelé à s'exprimer par référendum sur un texte dont le contenu réel reposerait sur une contradiction, sans doute délibérée, entre deux normes constitutionnelles opposées ? Dites-nous ce que vous voulez vraiment, monsieur le garde des sceaux ! Vous restez au milieu du gué. Si vous voulez rejeter dans les oubliettes de l'histoire la notion de développement durable, parce qu'elle est à vos yeux dépassée, assumez-le franchement et ne tergiversez plus ! Tranchez la question et ne laissez pas subsister un article 6 de la Charte de l'environnement orthogonal au texte que vous voulez faire adopter. Dites clairement ce que vous n'avez écrit qu'obscurément, à savoir que la garantie de préservation de l'environnement est plus importante, à vos yeux, que le développement économique et le progrès social, et que vous voulez donc faire prévaloir celle-ci sur ceux-là. Vous avez le droit d'avoir cette conviction. Nous ne la partageons pas. Cependant, pour la clarté du débat, il est essentiel de dire aux Français qu'il y a d'un côté ceux qui veulent inscrire la politique écologique dans le cadre du développement durable- nous en sommes ! -et ceux- vous en êtes ! -qui veulent l'en faire sortir. Vous avez raison de rappeler que le Conseil constitutionnel a l'habitude de concilier des principes constitutionnels dont les implications sont susceptibles C'est même le coeur de sa fonction, dans l'application de nos principes fondamentaux. Cependant, parmi nos droits fondamentaux, il n'existe pas de droits contradictoires, mais seulement des droits de nature différente, chacun avec leur limite fixée par la loi. Ils sont non pas antagonistes, mais relatifs,

à autrui ». Cela implique de concilier les droits des uns avec la liberté des autres, aucun droit n'étant absolu. L'article IV enfonce d'ailleurs le clou, pour ainsi dire : « L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance

à l'article 6 de la Charte de l'environnement, qui appelle une conciliation entre l'écologique, l'économique et le social. Certes, dans ce cas, le Conseil constitutionnel sait ce qu'il a à faire, directement guidé par l'énoncé même de nos principes fondamentaux : il ne s'érige pas en constituant délégué. Cependant, si on lui demande d'un côté de concilier l'écologique, l'économique et le social, puis, de l'autre, de garantir seulement l'écologique,

dans un passé lointain. Le Conseil constitutionnel ne peut pas, en effet, refuser de donner son plein effet utile à un texte adopté par le pouvoir constituant. Le choix sera binaire. Il n'y a pas de moyen terme entre le droit à la protection de l'environnement posé par la Charte, qui trouve sa limite dans les exigences du développement économique et du progrès social, et la garantie de la protection de l'environnement proposée par la Convention citoyenne, qui serait absolue, puisqu'aucune limite n'est énoncée pour en tempérer la portée. Telle est d'ailleurs sa seule raison d'être, malgré tous les efforts réalisés pour le dissimuler. En adoptant cette révision constitutionnelle dans les termes votés par l'Assemblée nationale, le Parlement et le peuple français se lieraient les mains. Ils signeraient un chèque en blanc au Conseil constitutionnel et aux groupes de pression susceptibles de le saisir. Ils contraindraient gravement les gouvernements et les législateurs de demain dans l'exercice même de la souveraineté nationale. aucune loi ne pourrait plus venir atténuer ou corriger la rigueur et la portée de mesures législatives déjà prises pour renforcer la protection de l'environnement. Le Président de la République, qui a engagé ce processus de révision constitutionnelle, devrait pourtant se souvenir que, lorsqu'il lui a fallu renoncer dans la précipitation à l'écotaxe, d'ailleurs votée contre la position du Sénat, il n'était finalement peut-être pas si inutile que le législateur ait eu alors la faculté constitutionnelle d'atténuer les contraintes excessives posées au nom de l'écologie, pour mettre fin Celui-ci a pu ainsi désamorcer la crise, en ajoutant la préoccupation économique et sociale à la préoccupation environnementale qui seule avait été prise en compte, à l'origine. Telle est la manière dont la Charte prévoit que le législateur pourra procéder. Or cette faculté, nous ne l'aurions plus demain, si les pouvoirs du Parlement devaient être drastiquement limités par un texte comme celui qui nous est présenté. C'est donc aussi en protecteur de nos institutions, de la fonction présidentielle et de la mission du Parlement que le Sénat doit rejeter la rédaction proposée par la Convention citoyenne pour le climat et souscrire à la proposition de notre commission des lois de réécrire le texte. Nous ne devons pas aliéner notre capacité souveraine de légiférer. Le Parlement ne doit pas se soumettre par avance aux aléas d'une jurisprudence constitutionnelle qui n'aurait pas été encadrée par l'expression claire de la volonté du constituant. Ce renoncement serait pour lui une véritable abdication. C'est au Gouvernement, ainsi qu'au Parlement, quand la loi est nécessaire, de déterminer librement la politique écologique de la Nation. Il leur appartient aussi d'en changer, si l'intérêt national et la volonté du peuple le commandent, sans que pèse sur eux l'épée de Damoclès d'un interdit invisible. La Constitution ne saurait prendre des gages sur les politiques de demain, qu'il s'agisse de l'environnement ou des autres domaines de l'action publique. doit pouvoir continuer à préférer la voie étroite, mais féconde, du développement durable à l'écologie de la décroissance que ce projet vise à inscrire dans le marbre de notre loi fondamentale. La discussion

revanche y avoir plusieurs politiques écologiques. Le Gouvernement avance masqué avec la sienne : il s'agit d'une politique écologique qui vise, grâce à une révision constitutionnelle, à rompre avec une conception du développement durable qui concilie écologie,

l'Assemblée nationale et le Gouvernement saisissent la main que nous leur tendons, en vue de parvenir à un accord sur cette base. Nous pensons que les Français sont profondément attachés au développement durable, qu'ils ne veulent ni d'une écologie punitive ni d'une écologie de la décroissance. Ils veulent à la fois le développement économique, celui de l'emploi, et le progrès social. Tel est le sens de cet amendement et de celui de la commission des lois.

110-1 du code de l'environnement. Afin de renforcer sa portée juridique et d'élargir son champ d'application, il doit être élevé au rang constitutionnel. Il faut lui conférer une valeur égale à celle des principes constitutionnels du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, généralement invoqués pour autoriser la mise sur le marché

Aussi, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande la consécration au rang constitutionnel du droit des générations actuelles et futures à vivre dans un environnement sain. Les nombreuses atteintes à la biodiversité et à l'environnement pourraient à terme entraîner la destruction de l'humanité. Ainsi, la France doit mettre en oeuvre toutes les politiques environnementales nécessaires, afin de limiter les effets de l'activité humaine à un niveau permettant à l'humanité de disposer des fonctions essentielles de la biosphère. Cette affirmation découle surtout d'un positionnement intergénérationnel. « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants

comptent parmi les menaces les plus imminentes et les plus graves qui pèsent sur le droit à la vie des générations actuelles et futures. » Nous souhaitons ainsi rappeler que nos décisions actuelles ont des conséquences sur la capacité des générations futures à vivre dans de bonnes conditions environnementales. Ce droit à un environnement sain, dans lequel il faut inclure le droit à l'eau, un air non pollué et les bénéfices de la biodiversité a été reconnu en France et inscrit dans la Charte de l'environnement de 2004. Il convient cependant d'en renforcer la portée juridique en l'érigeant en principe constitutionnel inscrit à l'article 1 de la Constitution. Quel

Ce concept a été proposé par une équipe internationale de vingt-six chercheurs, dont les travaux ont été publiés dès 2009. Il a d'ores et déjà été utilisé par de grands groupes industriels privés qui cherchent à confronter leur impact environnemental avec la capacité de notre planète à l'absorber.

Monsieur le rapporteur,

Cela justifierait, je crois- peut-être la réflexion pourrait-elle s'engager avec votre groupe, ma chère collègue -, que l'on prenne en compte, non seulement les limites planétaires, mais aussi les limites interstellaires ! S'agit-il d'un sous-amendement ?

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise le principe de non-régression. La gestion d'un avenir durable doit permettre de garantir que les acquis environnementaux ne seront pas remis en question. Le principe de non-régression protège les droits des générations futures, en renforçant l'exigence écologique lors des prises de décision.

Ce principe n'implique pas une impossibilité d'agir de la part des autorités. Il crée au contraire une obligation positive, notamment pour le législateur, de ne pas dégrader les avancées écologiques. Toutefois, en dépit de l'urgence climatique, certaines décisions législatives ou réglementaires sont moins-disantes au niveau environnemental : ce retour sur la protection de l'environnement et de la biodiversité est insupportable. Au vu des dernières décisions, qui ont permis au juge de valider un retour en arrière concernant la limitation des néonicotinoïdes, il est essentiel d'inscrire dans la Constitution que, à défaut de faire plus, on ne peut plus se permettre de faire moins.

constitutionnel consacre déjà le principe de non-régression. Dans une décision du 10 décembre dernier, le Conseil a ainsi dégagé de la Charte de l'environnement un principe de non-régression tempéré en matière environnementale. Il a considéré que le législateur « ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l'article 1 de la Charte de l'environnement. » Il a par ailleurs jugé que « les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. » Enfin, il a estimé que le législateur « doit prendre en compte,

une quasi-obligation de résultat, tantôt comme une obligation de moyens renforcée, et dont en réalité personne n'est capable de dire quelle est la portée juridique. Ce que nous souhaitons, vous l'aurez compris,

dans le cadre des principes du développement durable qui sont prévus par l'article 6 de la Charte de l'environnement. C'est pourquoi le groupe Les Républicains, dans son immense majorité, suivra la position du rapporteur François-Noël Buffet, que nous remercions Personne ne

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

nous entamons aujourd'hui l'examen en séance publique de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, afin de franchir, ensemble, une nouvelle étape dans la transformation et la réforme de notre dispositif de santé au travail. Je souhaite rappeler le choix réalisé par le Gouvernement, au début du mois de mars 2020, de proposer aux partenaires sociaux d'engager une négociation sur cet enjeu essentiel d'amélioration de la santé au travail. Les partenaires sociaux, après six mois de négociation, ont conclu un accord solide et équilibré

convergente en matière d'évolution de la santé au travail, après un travail approfondi, rendu encore plus essentiel en cette période de crise sanitaire. Le contenu de ces négociations est riche : développement de la prévention primaire, promotion de la qualité de vie au travail ou encore développement d'une offre de services en santé au travail efficace et adaptée auprès des entreprises et de leurs salariés. Nous aurons, je le sais, largement l'occasion d'y revenir dans les débats. Je me réjouis de la vitalité de notre dialogue social, qui, en cette période de crise, prend encore plus pleinement son sens. Nos partenaires sociaux ont su dépasser leurs antagonismes pour se faire force de proposition et concrétiser l'ambition d'une santé au travail résolument orientée vers la prévention. La démocratie parlementaire a ensuite pris très rapidement le relais, avec le dépôt, dès le 23 décembre 2020, de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, portée par les députés Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, et son adoption par l'Assemblée nationale en février dernier. Ce texte est désormais soumis à l'examen de votre assemblée. Cette nouvelle étape doit conforter l'existence d'une vision, partagée le plus largement possible, de la santé au travail dans notre pays. Je souhaite à cet égard souligner l'engagement et le travail de fond de chacun d'entre vous sur les questions de santé au travail, tout particulièrement celui de la commission des affaires sociales du Sénat, notamment

Cette forte implication doit permettre de donner corps à la négociation fructueuse des partenaires sociaux, en construisant le socle de sa traduction législative. Le Gouvernement se félicite de cette méthode de transposition- inédite, il est vrai -et veillera jusqu'à l'issue de la navette parlementaire à assurer le respect des équilibres obtenus par les organisations patronales et syndicales. Évidemment, la traduction de l'ANI du 10 décembre dernier ne se limite pas à un ensemble de mesures législatives. Un important chantier réglementaire, mais également organisationnel, est engagé, et les partenaires sociaux en sont bien logiquement des acteurs majeurs. Je souhaite d'ores et déjà valoriser certaines avancées inscrites dans cette proposition de loi, qui accélère la modernisation de notre système de santé au travail. n'en citerai que quelques-unes, puisque nous allons débattre du texte, à commencer par le renforcement de l'approche préventive de la santé au travail et de la traçabilité collective de l'exposition aux risques professionnels, notamment chimiques.

Je pense aussi à la création d'une procédure de certification de ces services, qui, associée à la tarification en plus complète transparence, permettra de soutenir leurs efforts de qualité sur l'ensemble du territoire.

des infirmiers et de la possibilité donnée, pour les infirmiers qualifiés, d'exercer en pratique avancée, ainsi que du développement des délégations de tâche. Votre commission, mesdames, messieurs les sénateurs, a effectué un travail important sur le texte adopté par l'Assemblée nationale, sans le dénaturer ni trahir les intentions de ses auteurs ou modifier les équilibres parfois délicats auxquels étaient parvenus les partenaires sociaux. Je souhaite souligner un point sur lequel la proposition de loi a subi une nette évolution lors de son passage en commission des affaires sociales au Sénat tenant compte des réalités de fonctionnement des petites entreprises, la commission a retenu que celles-ci pourraient définir leurs actions de prévention sans se voir imposer le formalisme d'un programme annuel de prévention.

les ajustements apportés sur le rendez-vous de liaison, pour permettre d'anticiper la reprise d'activité du salarié ; la définition d'un cadre pour la santé au travail des salariés des particuliers employeurs et des assistants maternels, qui, avec des avec des ajustements que je serai amené à proposer au cours du débat, me semble permettre d'instaurer, dans le cadre d'un dialogue social de branche, une prise en charge effective de ces publics. Parmi vos amendements de séance, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai noté de nombreuses propositions visant à préciser les missions des services de prévention et de santé au travail sur certaines thématiques ou certains publics spécifiques, parfois en les priorisant.

Comme j'ai eu l'occasion de le dire au cours de mon audition par votre commission des affaires sociales, j'ai également pu constater la forte mobilisation de ces services au cours de la crise sanitaire, mobilisation centrée actuellement sur la vaccination et l'accompagnement à la reprise et au retour progressif en entreprise. Le retour d'expérience de la pandémie doit permettre de construire, ensemble, un modèle de santé au travail plus proche de l'entreprise et des salariés, plus orienté vers l'accompagnement et le conseil pour la mise en place de mesures de prévention collective. me semble-t-il, sont prêts aux évolutions portées dans la proposition de loi. Il est en effet essentiel de moderniser notre système de santé au travail, pour qu'il puisse s'adapter et répondre aux enjeux des parcours professionnels du XXI siècle. Pour cette raison,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi fait suite à un long processus de démocratie sociale, ayant abouti à la conclusion

Cet accord a lui-même été précédé par la publication de plusieurs rapports proposant de faire évoluer notre système de santé au travail, dont celui que j'ai porté avec ma collègue Pascale Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, en 2019. Le diagnostic, largement partagé, est celui d'une grande hétérogénéité dans le contenu et la qualité de l'offre des services de santé au travail, qui sont confrontés à de multiples défis, dont celui de la démographie médicale, et d'une prévention primaire encore insuffisamment développée en entreprise. La proposition de loi se fixe ainsi pour premier objectif de consacrer le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, comme l'outil central dans la démarche de prévention et de traçabilité des expositions.

Nous concevons en effet le DUERP comme une protection, non seulement pour les travailleurs, mais également pour l'employeur. C'est notamment ce document qui lui permettra d'établir qu'il s'est bien engagé dans une véritable démarche de prévention. Soucieuse de tenir compte de la réalité des entreprises, notre commission a réservé l'élaboration d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail aux seules entreprises de plus de 50 salariés, comme vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire

L'évaluation des risques qu'elles conduiront débouchera alors sur la définition d'actions de prévention et de protection, dont la liste pourra être consignée dans le document unique. Afin de faire véritablement du DUERP un instrument de traçabilité des expositions collectives, objectif confirmé par l'ANI, notre commission a également veillé à réunir les conditions d'une conservation pérenne du document. Suivant un calendrier échelonné selon la taille des entreprises, le DUERP et ses mises à jour devront faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique centralisé et administré par les organisations patronales. Convaincue que l'établissement d'une frontière étanche entre la santé au travail et le reste du parcours de soins du travailleur n'a plus de sens à l'heure du concept ou « une seule santé », la commission a adopté plusieurs dispositions participant du décloisonnement de la santé au travail et de la santé publique. En complément de ses missions principales dans la prévention de l'altération de l'état de santé du travailleur du fait de son travail, elle a ainsi reconnu la contribution de la médecine du travail à l'atteinte d'objectifs de santé publique qui permettent, au cours de la vie professionnelle, de préserver un état de santé compatible avec le maintien en emploi. Si le dispositif du médecin praticien correspondant, préconisé par l'ANI, doit permettre aux SPST de faire appel aux médecins de ville pour renforcer leurs ressources médicales, nous considérons qu'il ne peut constituer une solution durable au problème de la démographie médicale. Afin de ne pas dénaturer la spécialité de la médecine du travail, dont la fine connaissance du milieu de l'entreprise est déterminante pour un suivi de qualité, la commission a donc encadré le recours au médecin praticien correspondant. Celui-ci sera limité aux situations dans lesquelles les ressources du SPST ne lui permettent pas d'assurer ses missions dans le respect des délais réglementaires. Pour répondre au défi de la démographie médicale, nous misons plutôt sur un renforcement de l'attractivité de la santé au travail, tant par la valorisation des compétences complémentaires acquises par les médecins du travail en prévention que par une montée en compétences cliniques et paracliniques des infirmiers, dont la contribution à la prévention mérite d'être reconnue et soutenue. Tel est, mes chers collègues, l'esprit dans lequel la commission des affaires sociales a abordé l'examen de ce texte. Elle vous demande en conséquence d'adopter cette proposition de loi, sous réserve de l'adoption de quelques amendements qui contribueront encore à l'enrichir. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce texte vise à répondre, à la suite de l'accord national interprofessionnel du du 9 décembre dernier, à un enjeu majeur : la promotion de la prévention primaire, au moment même où nous sortons à peine d'une culture de la réparation. Selon la dernière enquête du ministère du travail, moins de 40 % des entreprises employant moins de dix salariés ont élaboré ou actualisé au cours de l'année leur document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, qui est pourtant obligatoire. Pis encore, cette proportion est en baisse par rapport à la précédente enquête, qui portait sur l'année 2013. La proportion de TPE ayant mis en oeuvre des actions de prévention contre les risques physiques aurait ainsi diminué d'au moins 10 % entre 2013 et 2016. Le constat est donc sans appel : la culture de la prévention est très insuffisamment répandue au sein des TPE et PME, qui vivent encore la santé au travail comme un ensemble de contraintes administratives, et non comme un levier d'amélioration de leur performance. L'ambition de cette proposition de loi est précisément de systématiser la démarche d'évaluation des risques professionnels dans toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, et de garantir sa traduction opérationnelle dans la mise en oeuvre d'actions de prévention et de protection. À cet effet, les services de santé au travail, renommés « services de prévention et de santé au travail », devront jouer un rôle pivot dans l'accompagnement des employeurs, tout tout particulièrement auprès des TPE et PME. Or, en la matière, les partenaires sociaux se sont rejoints, dans le cadre

obligatoirement un ensemble socle de services, ainsi que, de manière facultative, une offre de services complémentaires qu'il déterminera. Soucieuse de garantir que les SPSTI proposeront à l'ensemble des entreprises adhérentes les prestations les plus homogènes possible, la commission a précisé la définition de cette offre socle. La proposition de loi revoit en conséquence, à l'article 9, les modalités de tarification des SPSTI. Le texte issu de l'Assemblée nationale confirme implicitement le principe jurisprudentiel du calcul de la cotisation en équivalents temps plein, ou ETP, qui est source de contentieux, peu respecté en pratique et ne correspond pas à la réalité des missions des SPSTI- en matière de prévention et de santé au travail, on ne peut effectuer un suivi partiel des salariés. La commission propose donc de consacrer un mode de calcul, et non proratisé en ETP. Par ailleurs, suivant le souhait des partenaires sociaux affirmé dans l'ANI, elle a inscrit dans le texte le principe d'un « tunnel » pour encadrer la fixation de la cotisation par référence au coût moyen national de l'ensemble socle de services. Le deuxième apport de la proposition de loi au sujet de la qualité et de l'effectivité des services rendus, également issu de l'ANI, est la mise en place d'une procédure de certification des SPSTI par un organisme indépendant et accrédité. Favorable à ce dispositif, la commission a souhaité que les partenaires sociaux aient l'initiative dans la définition du cahier des charges, le Comité national de prévention et de santé au travail, le CNPST. L'Assemblée nationale a par ailleurs élevé au niveau législatif la procédure d'agrément administratif à laquelle sont soumis tous les SPST, sans toutefois renforcer sa portée. La commission a introduit, en complément de cette procédure, un régime d'administration provisoire qui doit permettre, sans interrompre le service, de lui donner les moyens de se réorganiser lorsque sa gouvernance est défaillante. La proposition de loi franchit une première étape dans l'amélioration du suivi de l'état de santé de certaines catégories de travailleurs, suivi aujourd'hui insatisfaisant. Sont concernés, en particulier, les indépendants ou encore les intérimaires. Nous souscrivons à cet objectif, et la commission a enrichi le texte sur ce point, en ouvrant au chef d'entreprise la possibilité de bénéficier du suivi délivré par le SPST auquel adhère son entreprise et en proposant des modalités spécifiques de suivi des salariés du particulier employeur. Des améliorations pourront encore être apportées au texte lors de nos débats, avec l'objectif partagé de renforcer la prévention et le suivi de l'ensemble des travailleurs.

les rapporteurs, mes chers collègues, lors de la préparation de mon intervention, j'ai retrouvé une citation de Pierre Dac qui m'a semblé fort à propos pour notre débat de ce jour : « Le travail, c'est la santé ... mais à quoi sert alors la médecine du travail ? »

musculo-squelettiques, à l'exposition à des matières ou substances dangereuses ou encore aux risques psychosociaux. Longtemps passées sous silence, elles ont été identifiées, puis considérées progressivement. Le rôle de la médecine du travail est donc fondamental, notamment pour la détection, la prévention et la protection face à ces risques. Toutefois, la baisse du nombre de médecins du travail ne peut qu'affaiblir l'accompagnement que les travailleurs sont en droit d'exiger. De plus, notre paradigme se devait d'être réévalué, et le concept invite à un rapprochement entre le suivi dans le cadre du travail et la médecine de ville. Cela correspond à une évolution de nos sociétés vers une vie plus équilibrée et sans doute, nous l'espérons,

Depuis mon élection en tant que parlementaire, je milite pour une démocratie plus apaisée, qui écoute et sollicite les corps intermédiaires. Ces corps sont une source de propositions et d'informations essentielles pour le législateur. En étant au plus proche du terrain, dans les entreprises, ils nous communiquent régulièrement l'état des demandes, l'ambiance, les ressentis, mais aussi les difficultés vécues par les salariés, pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible. Quand je vois que cet accord national interprofessionnel a été signé par l'ensemble des organisations patronales et syndicales, à l'exception de la Confédération générale du travail, la CGT, et que nous sommes capables de le transformer en un texte ambitieux pour la santé des travailleurs, mon attachement au paritarisme et au dialogue social en sort renforcé. Le paritarisme n'est pas le concurrent de la démocratie parlementaire ; il est son indispensable complément ! Je tiens par ailleurs à féliciter nos rapporteurs Pascale Gruny et Stéphane Artano

savoir déceler les premiers signaux d'un mal-être au travail peut sauver une carrière et permettre à un salarié de se remettre sur les rails. Cette prévention doit être la même partout, et je me réjouis que ce texte mette fin aux inégalités que l'on peut observer entre les entreprises en fonction de leur taille ou de l'engagement de leurs dirigeants sur ces questions essentielles. Cette prévention s'accompagne d'une simplification bienvenue des procédures. J'entends effectivement les patrons de nos TPE et PME qui, loin de ne pas être sensibilisés à la santé de leurs salariés, se plaignent régulièrement de procédures trop complexes, trop techniques ou trop nombreuses, la prévention est le talon d'Achille du système de santé français. Un autre point essentiel de ce texte est la reconnaissance de la contribution de la santé au travail à la santé publique. « Enfin ! Je ne sais pas pourquoi, mes chers collègues, nous avons si longtemps mis une barrière entre la santé publique et la santé au travail. Comme si nous revenions chez nous dans un autre corps que le nôtre ou que nous étions capables de laisser sur le pas de notre porte tous nos tracas professionnels. C'est évidemment faux, chacun le sait ici. C'est pourquoi je salue pleinement la dynamique engagée par nos rapporteurs. La santé au travail, au même titre que la santé maternelle ou infantile, la santé environnementale, la santé le sport, etc. a toute sa place dans la réalisation des objectifs de notre politique nationale de santé publique. C'est sans doute évident pour certains, mais cela va mieux en le disant : la santé publique peut et doit concerner tous les domaines de la santé.

que les partenaires sociaux se sont accordés sur le diagnostic d'une « grande hétérogénéité » des prestations rendues par les SPST, notamment en matière de prévention, je trouve cela tout simplement insupportable. Or c'est dans ce domaine que l'attente est la plus forte de la part des employeurs et des salariés. Nous devons nous engager pour que chaque salarié dispose de la prévention en santé au travail dont il a besoin. Ce texte permettra, je l'espère, et nous devrons y veiller particulièrement, de combler les trous dans la raquette et de s'assurer que les salariés disposent d'un socle minimal ambitieux. Un troisième axe développé dans cette proposition de loi m'a aussi particulièrement interpellé. Il met en lumière la désinsertion professionnelle- le terme est peut-être

: création d'une cellule pluridisciplinaire dédiée ; systématisation des échanges d'informations entre les organismes d'assurance maladie et les services concernés ; mise en place d'une visite à mi-carrière ; organisation de visite de préreprise et reprise, ainsi que de rendez-vous de liaison avec l'employeur. Ces mesures vont dans le bon sens. Enfin, le quatrième et dernier sujet important aux yeux de mon groupe est la revalorisation de l'engagement des professionnels de santé au travail. Les inégalités d'accès aux ressources médicales en santé sur notre territoire sont un véritable problème. Face à la pénurie médicale à laquelle nous sommes confrontés,

porte une proposition ambitieuse pour les travailleurs de notre pays et pour leur santé. J'espère qu'elle est la première d'un cycle de propositions de loi importantes, coconstruites et pragmatiques, que nous pourrons nous féliciter d'adopter. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, chaque année, on ne déplore pas moins de 50 à 600 morts au travail, plus de 30 000 incapacités permanentes et plus de 600 000 arrêts de travail. L'ampleur de ces chiffres révèle l'importance du sujet de la santé et du bien-être au travail de nos concitoyens. La crise du covid-19 et les périodes de confinement successives ont entraîné une dégradation de la santé des travailleurs, avec une hausse importante des troubles psychosociaux. Cette crise a également montré toute l'importance du médecin du travail, relais des pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie au sein de l'entreprise et interlocuteur privilégié des salariés en télétravail. Dares, au début de l'année 2021, l'état de santé psychique des travailleurs s'est fortement dégradé, avec un doublement du risque de dépression et une forte détérioration de la santé perçue, et cela d'autant plus que leurs conditions de travail ont été affectées par la crise sanitaire. Les actifs sont également plus nombreux à déclarer des troubles du sommeil, des douleurs plus fréquentes ou plus fortes. Le texte que nous examinons aujourd'hui a pour ambition de réformer l'offre de services et la gouvernance des services de santé, ainsi qu'à améliorer le suivi médical des salariés et la prévention

il passe à côté d'enjeux essentiels en matière de santé au travail, surtout en ce qui concerne la prévention primaire des risques professionnels ; il provoque même une confusion entre la santé au travail au regard de l'organisation du travail- les critères de pénibilité ont par exemple disparu -et la santé du travailleur en entreprise, en faisant la promotion individuelle de la santé- consommation de tabac ou d'alcool, pratique De même, le texte ne contient aucun apport concernant la reconnaissance des maladies professionnelles, en particulier celles qui sont liées aux risques psychosociaux. Ces derniers constituent pourtant le deuxième groupe de pathologies les plus fréquentes dans le monde du travail, après les troubles musculo-squelettiques. Au-delà de ces insuffisances, ce texte comporte certains risques pour les travailleurs, en ce qu'il organise une certaine déresponsabilisation de l'employeur en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés. De nombreuses mesures tendent à transférer cette responsabilité vers les salariés eux-mêmes ou vers les services de prévention et de santé au travail. L'instauration d'un passeport prévention à l'article 3 en est la parfaite illustration. Ce passeport semble être un blanc-seing permettant aux employeurs de se dégager de leur responsabilité en matière de sécurité, au motif qu'un travailleur a été préalablement formé. formé. Un autre point doit retenir notre attention : la possibilité pour le médecin du travail d'accéder au dossier médical partagé, le DMP. Si donner accès à ce dossier au médecin du travail pour y verser des éléments présente un intérêt indéniable, l'inverse n'est pas vrai les données personnelles de santé des salariés ne doivent pas être visibles par le médecin du travail ! En effet, la possibilité pour le médecin du travail d'accéder à ces données, même avec l'accord du patient, risque d'être préjudiciable aux salariés, en particulier lors des visites d'embauche et de reprise du travail, surtout lorsqu'il y a une nécessité d'adaptation à l'emploi. Enfin, ce texte ne répond pas au problème concret de la pénurie de médecins du travail. Nous comptons aujourd'hui 1 médecin pour 4 000 salariés : c'est deux fois moins qu'il y a quinze Pour faire face à cette pénurie, vous proposez de recourir à des médecins correspondants. C'est pour le moins surprenant, compte tenu du contexte de désertification médicale que connaît actuellement notre pays. En outre, ces médecins correspondants, même avec deux années de formation complémentaires, ne pourront pas faire de la prévention en entreprise- c'est pourtant le rôle essentiel du médecin du travail. sanitaire, comme dans un grand nombre d'autres domaines, a mis en lumière d'importants dysfonctionnements : pénurie de médecins du travail, systèmes illisibles et difficiles d'accès, inégalités territoriales. de loi, porteuse de grands espoirs, n'apporte en réalité aucune solution concrète, et nous le regrettons. Ainsi, en l'absence d'amélioration significative du texte à l'issue de nos débats, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne votera pas cette proposition de loi.

présente proposition de loi est la transcription. Celle-ci prévoit une réforme de la santé au travail visant à harmoniser et à renforcer les actions de prévention des risques professionnels. L'article 1 formalise ce changement de paradigme en renommant les services de santé au travail en services de prévention et de santé au travail ; il s'agit de structures financées par les cotisations des entreprises. Les consultations d'un médecin du travail sont très variées, allant des conseils de prévention à la reconnaissance d'inaptitudes médicales au travail, ce qui entraîne de nombreux mécontentements de la part des salariés ou de l'entreprise,

Le médecin du travail partage son temps entre les visites médicales, les tâches administratives et les actions en milieu de travail. Il consacre un temps essentiel à l'étude des postes et à l'analyse des risques au sein des entreprises qu'il visite.

Il est également compétent en matière de rangement des produits nocifs et dispense ses conseils sur la structure et l'organisation même de l'entreprise. Il a donc, par nature, un rôle de prévention fondamental concernant aussi bien les risques chimiques et physiques que le suivi à long terme des personnes exposées. Sous la responsabilité de l'employeur, il participe à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels identifiés dans l'entreprise. Véritable carte d'identité de l'entreprise, ce document est le point de départ des actions de prévention nécessitant une mise à jour annuelle. Un amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à étendre la durée de conservation du document à quarante ans au minimum, ce qui permet de tenir compte d'effets nocifs sur la santé à très long terme.

des services de prévention et de santé au travail. La commission des affaires sociales du Sénat a d'ailleurs étendu ce suivi aux chefs d'entreprise. La création d'un médecin praticien correspondant, formé en médecine du travail, contribuera à pallier la pénurie de médecins du travail dans les territoires concernés. Certaines missions pourront en outre être déléguées aux infirmiers qualifiés, sous la responsabilité du médecin du travail.

et de la prévention des maladies professionnelles. La complémentarité de leurs activités doit être renforcée. Le médecin du travail n'est pas l'acteur du suivi personnalisé d'un traitement- aux bêtabloquants, par exemple -, ni de l'adaptation de ce traitement.

entre les organismes de sécurité sociale et les services de prévention et de santé au travail. L'accord du patient est essentiel, c'est un point sur lequel nous devons rester extrêmement vigilants. Pour autant, c'est aussi une évolution que l'on peut espérer dans un certain nombre de situations.

prenant la mesure des responsabilités régaliennes sur la prévention de la santé des travailleurs. C'est d'autant plus vrai que, en France, un écart de presque dix ans d'espérance de vie en bonne santé sépare l'ouvrier du cadre, et cela en grande partie du fait du travail. Vous auriez dû inviter les parlementaires à un véritable travail et à un débat de fond. Mais vous les en avez privés par vos ordonnances de 2017, dont je veux rappeler ici une mesure inique

altérant la santé ont ainsi été retirés ! De plus, c'est dénier au législateur le principe que, en matière de santé et de sécurité au travail, tout ne se négocie pas. Derrière les statistiques, il y a des accidents du travail- plus de 500 morts sont comptabilisées chaque année dans le secteur privé -, des maladies professionnelles et des inaptitudes. Nous ne pouvons être totalement tenus par l'accord de compromis signé dans le cas d'un équilibre des forces sociales ; vous conviendrez en effet que celui-ci reste en défaveur des salariés.

l'effacement du médecin du travail. C'est une tendance ancienne, car, malgré les alertes, rien n'a été entrepris pour lutter contre les sous-effectifs ou pour renforcer l'attractivité, y compris pour les médecins collaborateurs. Force est de constater l'inaction pour contrer la baisse des seuls professionnels protégés. Nous nous élevons notamment contre l'introduction des médecins praticiens correspondants. Rarement les médecins du travail, dont la spécialisation dure quatre ans, n'ont fait l'objet d'une telle dépréciation, voire d'un tel mépris. Cela explique que l'attractivité soit en berne. Au-delà, c'est bien le lien entre santé et travail, pour prévenir à la source toute altération de la santé par le travail, qui est nié.

Elle trouve ses racines dans la loi Villermé de 1841. Depuis lors, le cadre législatif l'encadrant n'a cessé de croître, afin de protéger davantage les salariés ; je pense notamment à la loi du 9 avril 1898 prévoyait l'indemnité des salariés en cas d'accident survenu au travail. Quant aux lois de 2002, de 2011 et de 2016, elles furent autant d'étapes renforçant le droit à une protection de la santé au travail. d'un service de santé au travail interentreprises, ou SSTI. On estime à 7 millions le nombre de visites réalisées chaque année. Mais les médecins du travail et les collaborateurs médecins ont perdu près de 10 % de leurs effectifs entre 2015 et 2019.

Aussi, de la stratégie nationale de santé 2018-2022 mise en place par le Gouvernement aux réflexions menées par l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, en passant par les rapports parlementaires, nombreux sont les travaux qui ont clairement identifié les problématiques de ce système ces dernières années. Les rapporteurs de ce texte, ici, au Sénat, ont rédigé un rapport proposant des évolutions destinées à garantir un service universel de la santé au travail de qualité pour tous les travailleurs. proposition de loi, à l'Assemblée nationale, se sont quant à eux penchés sur la manière de moderniser la santé au travail en France, la rénovation de sa gouvernance. Je me réjouis que les parlementaires se saisissent d'un sujet plus que jamais déterminant, à la faveur de la crise sanitaire. Leurs travaux auront, entre autres, permis d'alimenter les réflexions des partenaires sociaux qui, dans l'ANI, ont repris plusieurs des propositions formulées. il aura fallu de longues discussions et de nombreuses négociations avant de parvenir, le 9 décembre 2020, à la conclusion de l'ANI pour une prévention pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail, signé par la quasi-totalité des partenaires sociaux, excepté la CGT. la CGT. Mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est le fruit d'un long processus de démocratie sociale et parlementaire et, à l'instar des députés, il nous faut veiller à ce que la transcription de l'ANI dans la loi respecte aussi bien son contenu que son équilibre. La proposition de loi s'articule autour de quatre axes. Premièrement, renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail. Deuxièmement, améliorer la qualité du service rendu par les SST. Troisièmement, Troisièmement, renforcer l'accompagnement de certains publics, notamment vulnérables, et lutter contre la désinsertion professionnelle. Quatrièmement, et enfin, réorganiser la gouvernance de la santé au travail, que celle-ci soit interne aux SST ou concerne le pilotage national et territorial de celle-ci.

La commission des affaires sociales, saisie au fond, s'est réunie le mercredi 23 juin 2021 pour examiner le rapport de nos collègues Stéphane Artano et Pascale Gruny- je loue le travail d'enrichissement qu'ils ont fourni. Bien que la commission partage les principaux objectifs de la proposition de loi, elle a veillé à garantir le caractère opérationnel de plusieurs de ses dispositions phares et à réunir les conditions d'un développement effectif de la prévention au sein des entreprises. précisé la définition de l'offre socle de services proposée par les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les SPSTI ; elle a réaffirmé le rôle du médecin du travail dans l'animation et la coordination d'une équipe pluridisciplinaire, qui a vocation à se diversifier se diversifier ; elle a étendu aux services de prévention et de santé au travail des obligations de mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité, en faveur d'une meilleure protection et d'une exploitation plus efficace des données en santé au travail.

Enfin, nous entendons nous assurer du rôle central des acteurs de la santé au travail au sein des conseils locaux de santé mentale, dont nous savons l'importance. Mes chers collègues, la transcription dans la loi de l'ANI respecte aussi bien son contenu que son équilibre. Concours de circonstances, elle intervient au moment où la Commission européenne a publié, il y a quelques jours, le cadre stratégique qui viendra orienter sa politique en matière de santé et de sécurité au travail.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi visant à renforcer la prévention en santé au travail transcrit dans la loi l'ANI signé le 10 décembre 2020 par le patronat et par une partie des organisations syndicales de salariés. Cet accord sur de nouvelles mesures pour la santé au travail est déconnecté de la réalité de la situation des travailleuses et des travailleurs. Alors que la crise sanitaire a profondément bouleversé les organisations de travail, le texte ne prévoit aucune mesure sur l'encadrement du recours au télétravail.

profond recul pour les représentants du personnel et pour la santé et la sécurité des travailleurs- la pandémie a pourtant montré combien ils étaient essentiels. Ce texte ne prévoit rien sur la mise en place d'une véritable politique de prévention primaire des risques professionnels prenant en compte la pénibilité des postes et l'usure professionnelle. En réalité, la proposition de loi ne s'attaque qu'à une partie extrêmement réduite de la santé au travail. De nombreux sujets ne sont pas abordés, tels que la prise en compte de la pénibilité, la question du temps de travail, du travail de nuit et de la prévention des violences sexistes et sexuelles, ou encore la multiplication des licenciements pour inaptitude au poste de travail.

; elle crée un passeport prévention, mais celui-ci renvoie la responsabilité de la santé et de la sécurité sur chaque salarié, sans prendre en compte le travail réel et son organisation. En outre, le texte introduit un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, qui remet en cause la visite de préreprise en court-circuitant le médecin du travail. Ces rendez-vous sont pourtant fondamentaux dans la prévention des inaptitudes et permettent d'éviter les pressions managériales. Face à la pénurie de médecins du travail, le Gouvernement a choisi de créer des médecins praticiens correspondants et de déléguer les fonctions et les missions du médecin du travail aux infirmières. Nous pensons, au contraire, que la situation exige d'augmenter le nombre de places au concours des médecins du travail, à revaloriser la formation dans les universités et à améliorer les conditions de travail. La logique de rationalisation de la santé au travail justifie l'instauration d'une certification des services de prévention par des organismes privés, qui remplissent pourtant une mission de service public.

Les garanties ne sont pas suffisantes pour nous rassurer. En effet, si l'accord exprès du salarié est prévu, comment allez-vous garantir l'absence de pression sur les salariés ou vous assurer que ce choix a été fait de manière éclairée ? Le texte prévoit l'archivage du document unique d'évaluation des risques pour une durée minimum de quarante La commission des affaires sociales a prévu la création d'un site internet pour l'archivage, géré par les organisations patronales. Pour notre part, nous considérons que la traçabilité

En conclusion, le texte ne prévoit aucune proposition pour de véritables droits pour les salariés et leurs représentants. Pourtant, les syndicats et les professionnels de la santé au travail en formulent : amélioration du suivi des salariés privés d'emploi, allongement des délais de contestation des avis d'inaptitude, rattachement des SST au travail à la sécurité sociale, rétablissement des CHSCT. Enfin, mes chers collègues, je tenais à évoquer un point concernant nos travaux et notre rôle en tant que parlementaires. Un grand nombre d'amendements ont été déclarés irrecevables sur le fondement de l'article 45 de la Constitution : 44 amendements que nous avions déposés ne seront donc pas étudiés, ont été considérés comme des cavaliers législatifs. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera contre cette proposition de loi, qui passe à côté des enjeux essentiels de la santé au travail

Voilà déjà une bonne nouvelle ! Ce n'est pas la première fois que notre assemblée examine un texte visant à transposer un accord national interprofessionnel,

Nous réformons donc notre droit du travail après que les partenaires sociaux se sont mis d'accord : c'est la concrétisation des jalons posés par la loi Larcher en 2007 pour moderniser les règles afférentes au dialogue social, texte dont j'avais eu l'honneur d'être le rapporteur au Sénat. Le sujet de cette après-midi est d'actualité. Les précédents orateurs l'ont rappelé : nous avons vu tout au long de la crise sanitaire que le traitement curatif des risques professionnels ne suffit pas. Il convient de renforcer la vigilance en amont et de mieux identifier les risques, notamment psychosociaux, susceptibles de toucher les salariés.

La proposition de loi soumise à notre examen comporte des avancées significatives. Elle élargit notamment le champ de la prévention à la désinsertion professionnelle, qui contribue à des situations de chômage de longue durée et d'éloignement du marché du travail préjudiciables

je pense à l'amélioration du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, qui représente une étape importante, et à l'instauration d'un passeport prévention, souhaité par les signataires de l'ANI.

La clarification des services que les SPST sont tenus d'offrir aux salariés est la bienvenue. En parallèle, le déploiement d'une offre socle ne pourra que renforcer l'égalité entre les différents services oeuvrant à l'échelle nationale. L'ANI consacrait des dispositions spécifiques à de nouvelles catégories de travailleurs, notamment les personnes en situation de handicap et les salariés d'entreprises sous-traitantes. texte reprend ces diverses dispositions de bon sens, qui permettront une couverture plus large des risques professionnels. De plus, je note que les dispositions concernant la réorganisation de la gouvernance des services de prévention

simplifie la visite de mi-carrière en la rapprochant des dispositifs existants. Sensible aux fractures territoriales et aux risques de désertification médicale,

À ces méthodes de travail, nous préférons de loin celles de la démocratie sociale et de la négociation syndicale, qui aboutissent à des compromis exigeants, mais réalistes. Vous l'avez compris : les élus du groupe Les Républicains accueillent ce texte avec un esprit constructif et fidèle aux équilibres trouvés par les partenaires sociaux. L'Assemblée nationale est parfois sortie de ce cadre, contrairement à nos rapporteurs, Pascale Gruny et Stéphane Artano, qui sont restés plus fidèles à l'accord négocié, tout en l'améliorant.

Assurer la santé des ouvriers ou des salariés est une préoccupation ancienne : il y a 2 500 ans, on en parlait déjà sur les chantiers pharaoniques. Plus près de nous, Hippocrate identifia le plomb comme cause des maladies des ouvriers métallurgistes.

Son évolution vers une approche de prévention des risques professionnels et de santé au travail, tant physiques que psychologiques, s'amorce avec les lois Auroux de 1982, créant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

Le volet dédié à la gouvernance de ces services garantit le partage des informations médicales, y compris entre l'assurance maladie et les services de prévention au travail. La représentation des salariés n'est pas oubliée, et l'effort doit se poursuivre pour que les représentants des salariés des petites et moyennes entreprises

L'article 14 contribue au maintien dans l'emploi des personnes malades ou handicapées. Quant à l'article 16, instaurant une visite de mi-carrière, il représente une véritable avancée. Je suis favorable à ces dispositifs, qui inscrivent la santé au travail dans une logique pluridisciplinaire plus ouverte sur la médecine de ville, associant les psychologues, les kinésithérapeutes, les ergonomes et bien d'autres

La pandémie de la covid-19 a mis en exergue l'importance du volet de prévention en santé au travail. Les employeurs et les partenaires sociaux ont dû déployer dans l'urgence les moyens d'assurer la sécurité des salariés face à la contamination virale, que ce soit en favorisant le télétravail ou en fournissant des matériels de désinfection et de protection. En parallèle, d'autres défis se profilent, avec l'émergence de nouveaux types d'emplois

Pour répondre à ces défis, la santé au travail devra reposer sur une approche et des équipes pluridisciplinaires, mieux à même de redonner la santé aux salariés. Le présent texte nous semble contribuer à cette évolution, et les élus du groupe du RDSE le voteront, même si la problématique de la démographie médicale demeure préoccupante ! La parole

: il s'agit de transformer un système de santé au travail jugé unanimement à bout de souffle- manque de médecins du travail, coordination insuffisante des multiples acteurs, couverture imparfaite des besoins des petites et moyennes entreprises, des travailleurs indépendants, des salariés multi-employeurs ou des salariés portés. La création d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises est porteuse d'espoir pour les salariés comme pour les employeurs. Cette structure est constituée d'un panel représentatif des différents intervenants de ces services. Toutefois, les parties prenantes ne seront pas en mesure d'identifier une problématique commune à partir d'un ensemble de situations individuelles similaires relevées.

Néanmoins, cette mesure pourrait aller plus loin ; de nombreux salariés en situation de handicap ne demandent pas leur reconnaissance comme travailleurs handicapés. Or le référent handicap devrait pouvoir informer l'ensemble des salariés des droits spécifiques des personnes handicapées et de l'intérêt de ce statut.

L'article 15 de cette proposition de loi autorise les professionnels de santé à recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance pour le suivi de l'état de santé des travailleurs. Si la pandémie a démontré l'utilité du recours à la téléconsultation, la présence physique du salarié et du médecin au rendez-vous médical doit rester le principe, la téléconsultation ayant valeur d'exception. La loi doit fixer cette règle. S'agissant des assistants maternels, nous avons défendu en commission des amendements visant à ouvrir la possibilité d'un accord de branche étendu afin d'élaborer des mesures spécifiquement adaptées à ces métiers.

En conclusion, malgré quelques avancées, ce texte se démarque par ses nombreuses lacunes. Il n'évoque pas le lien avec l'inspection du travail ; il n'aborde ni la question de la responsabilité des employeurs en cas d'accident du travail ou de suicide, ni la pénibilité, ni la qualité de vie au travail ni la santé des travailleurs en inter-contrat

l'encadrement du télétravail, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre des plans de prévention, de la mise en place d'un cadastre des maladies professionnelles, des procédures de contestation des avis d'inaptitude ou encore de la suppression des CHSCT- ma liste n'est pas exhaustive. Ces sujets sont directement en lien avec la thématique de cette proposition de loi.

Je centrerai mon propos sur ce second point. Certains d'entre nous, qui siégeaient déjà dans cet hémicycle en 2012, se souviennent des débats menés pour élaborer une définition pénale du harcèlement sexuel. Sans en retracer l'historique, rappelons que cette définition

J'ai été alertée par plusieurs associations, dont l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l'AVFT, et par diverses organisations syndicales qui montrent très bien le danger d'une telle harmonisation. Actuellement, si les conseils des prud'hommes et les chambres sociales des cours d'appel peuvent rendre des jugements de licenciement de harceleurs, c'est précisément parce que les définitions ne sont pas identiques : en droit du travail, il n'y a pas à démontrer de quelle manière les agissements ont été imposés à la victime. Cette distinction et fondamentale justifiée : au pénal, il est nécessaire de démontrer l'élément moral de l'infraction, alors qu'en droit du travail le juge se contente de la matérialité des faits.

Mme Cohen : dans le code du travail, l'élément intentionnel du comportement de l'auteur n'est pas mentionné. Cet amendement, soutenu par les organisations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes,

Sur ce sujet important, faire preuve de précision rédactionnelle est bien évidemment indispensable. Il nous semble que cette modification serait cohérente avec la rédaction des dispositions actuelles du code du travail. Le Conseil d'État, dans son avis sur cette s'est prononcé en faveur d'une harmonisation entre les deux codes. Cependant, de notre point de vue, cette nécessaire harmonisation n'est pas incompatible avec le maintien des spécificités du droit du travail, qui se révèlent plus protectrices des victimes. En conséquence, la commission a émis un avis favorable

Mme Raymonde Poncet Monge. La sécurité au travail est une liberté fondamentale, bafouée quotidiennement par des manquements qui entraînent parfois des accidents, des mutilations, des handicaps, des incapacités de travail, ou même la mort dans les cas les plus extrêmes. Depuis des années, les pouvoirs publics n'arrivent plus à faire reculer le taux d'accidentalité. Au contraire, dans certains secteurs, on assiste

et de renforcer la sanction en cas de manquement par une indemnité minimale équivalente à trois mois de salaire. Quel

entre code du travail et code pénal, comme il est prévu à l'article 1. Il convient ainsi de préciser, parmi les missions des services de prévention et de santé au travail, que la lutte contre le harcèlement sexuel doit être associée aux violences « sexistes ». Aucune décorrélation ne peut être envisagée. Quel est l'avis de la ? La notion de harcèlement sexiste, que cet amendement tend à mentionner au titre des missions des services de santé au travail, n'a pas vraiment de définition juridique.

pour ne pas aborder ce problème de fond et, ainsi, ne pas remettre en cause des pratiques répandues, usuelles, mais inacceptables. Si notre amendement tend à prévoir des sanctions pour rappeler les employeurs à leurs manquements, ce qui est nécessaire et permettra aussi de combler un vide juridique, nous regrettons de ne pouvoir agir en amont en proposant des plans spécifiques de prévention obligatoires et surtout des actions concrètes. J'en profite pour me réjouir que la ratification de la convention n° 190 de

Cette convention est historique et extrêmement ambitieuse. Considérer que notre droit actuel est suffisant pour la décliner et l'appliquer est une erreur. Il est dommageable que le Gouvernement, une fois de plus, se contente d'affichage, plutôt que de saisir cette occasion pour aller plus loin et vraiment protéger les femmes sur leur lieu de travail. Monsieur le secrétaire d'État, j'espère que vous entendrez ma requête, très largement partagée par toutes celles et tous ceux qui luttent contre les violences faites aux femmes. Il est encore temps de modifier le texte. En attendant,